Daniel Salmon, pour explication de vote.

article dispose : « En tout état de cause, ces travaux ne sont pas assimilables à la destruction de haie au sens de l’article L. 412 24. » Or cette rédaction ne permet pas à elle seule de couvrir toutes les méthodes de destruction. Ainsi, elle couvre les coupes de prélèvement pour récolter la biomasse, mais pas les destructions d’après coupe, avec broyage ou abroutissement des repousses, qui empêchent la haie de repartir. C’est tout sauf une gestion durable.

est à Mme la ministre. Cet amendement a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d’État la fixation des délais de réponse de l’administration

Madame la ministre, je vous remercie pour s’opposer à la destruction projetée ; d’autre part, le délai dans lequel elle peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique. Pourquoi est ce nécessaire ? Parce que ces délais doivent être cohérents avec les différentes procédures légales dont relève le régime unique de la

! Soyons plus clairs, soyons plus rapides, soyons plus réactifs. C’est d’ailleurs exactement ce que l’on demande tous les jours aux agriculteurs

Or, au vu de l’encombrement actuel de l’administration, une telle disposition pourrait revenir à laisser le champ ouvert à des autorisations multiples, faute de réponse, et donc à des destructions en masse. Ce risque est d’autant plus réel

Lorsque l’agriculteur dépose sa demande de destruction de haie, il ne sait pas si elle sera qualifiée de demande d’autorisation. Il serait préjudiciable qu’une absence de réponse à une déclaration du fait d’un retard de l’administration vaille acceptation, alors que le projet pourrait être en définitive soumis à autorisation.

et constitue un risque, eu égard aux enjeux attachés à la préservation des haies. D’une manière globale, convenons que l’arrachage d’une haie peut s’anticiper

applicables au fait de détruire une haie sans avoir obtenu une absence d’opposition, ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition.

« fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au I, sans avoir obtenu cette autorisation unique ». Oui !

La plupart des actes de classement en réserve naturelle interdisent, par principe, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés. La destruction de haies sauvages n’est donc pas juridiquement possible dans ces réserves. Quant aux haies composées de végétaux cultivés, on pourrait considérer qu’elles sont soumises à l’objectif de bon état de conservation du patrimoine naturel de la réserve naturelle, et qu’il n’est, partant, pas possible d’y porter atteinte.

Cet amendement vise à compléter l’alinéa 41, relatif aux mesures de prescription nécessaires en cas de destruction d’une haie. Il s’agit d’apporter la précision suivante : la possibilité ouverte à l’autorité administrative de fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts de la haie, tels qu’énoncés au nouvel article L. 412 24, vaut également lorsqu’il s’agit de la qualité de l’eau.

également préciser qu’il existe plusieurs coefficients par département, notamment pour tenir compte de la typologie des haies et de la valeur écologique de ces

Jean François Longeot. Le nouveau régime de protection et de mise en œuvre des plans de gestion durable des haies, créé par l’article 14 du présent texte, est censé s’appliquer aux haies situées sur les emprises des infrastructures linéaires et qui n’engagent pas leur gabarit de sécurité.

Pour s’assurer du bon respect de l’application de la loi et se donner les moyens d’atteindre l’objectif de replanter 50 000 kilomètres de haies d’ici à 2030, il semble en effet indispensable de disposer d’outils de suivi et de contrôle de ce type. Quel

et un coefficient de compensation en cas de destruction. Cet arrêté doit être pris après avis des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux.

est à Mme la ministre. Le Gouvernement propose de renvoyer à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) le soin de rendre un avis sur le projet d’arrêté préfectoral définissant les périodes d’interdiction de travaux sur les haies,

en mobilisant des compétences diverses, telles que celles des représentants de l’État, des élus locaux, des agriculteurs, ainsi que des associations.

d’aller au delà ni de multiplier les dates d’interdiction au sein d’un même département. Cela risquerait de créer une confusion en matière de règles applicables et de nuire aux objectifs de sécurisation des gestionnaires et propriétaires de haies et de simplification administrative.

d’informer l’acquéreur ou le preneur à bail de la présence de protections applicables aux haies lors de la mutation ou du changement des parties d’un bail rural n’est pas de nature à encourager la cession ou la mise à bail.

la proposition de loi en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie de notre collègue Daniel Salmon. Cette proposition de loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat la semaine dernière, repose sur une certification garantie par l’État pour valoriser la gestion durable des haies, développer les objectifs de valorisation énergétique du bois bocager et instituer une stratégie en faveur de la reconquête de la haie, afin de donner une assise législative au pacte en faveur de la haie, présenté fin 2023.

? Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas au Sénat ! La semaine dernière, monsieur Salmon, vous êtes parvenu à faire adopter à l’unanimité un texte magnifiant la haie et exaltant sa défense ; aujourd’hui,, nous avons assisté à plusieurs reprises à

vous présente donc de nouveau, mes chers collègues, un amendement d’appel qui vise à promouvoir les paiements pour services environnementaux. L’agriculture française, dans la variété de ses terroirs et des techniques employées, contribue à répondre aux besoins divers de la société. Au delà de sa fonction nourricière première, elle produit des externalités qui affectent positivement l’environnement, les paysages et la biodiversité, tout en permettant à tous les Français de profiter d’espaces valorisés et protégés

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

l’allégement des charges, la hausse des rendements et la juste rémunération –, je ne dis pas que la question de la valorisation des externalités positives sera secondaire, mais nous aurons déjà parcouru un sacré bout de chemin.

l’article L. 341 2 du code forestier précise que « ne constituent pas un défrichement », et ne sont donc pas soumises à autorisation, « les opérations ayant pour but de remettre en valeur » d’anciennes terres

forestier, vous le remarquerez, ne fixe pas de limite d’âge des peuplements. De surcroît, ce même article précise que « le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé

l’autonomie fourragère et ont donc besoin de prairies, lesquelles, je le rappelle, sont d’aussi bons capteurs de carbone que les forêts.

C’est une injustice profonde, fondamentale ! Eh oui ! Si nous n’arrivons pas à regagner de la surface agricole utile, nous ne progresserons pas en matière de souveraineté alimentaire. Il ne s’agit pas de s’attaquer à la forêt.

s’il le souhaite, il en aura la possibilité légale. C’est tout de même intéressant.

Il existe déjà un délit pour sanctionner les propriétaires défaillants. Malheureusement, je vous l’accorde, ces procédures sont lourdes et n’aboutissent pas toujours. Pour remédier à ce problème, le Gouvernement a défendu un amendement dans le cadre

! La difficulté à trouver un logement en bon état, peu coûteux, peu énergivore et proche de l’exploitation freine de nombreux candidats à l’installation, en particulier les « non issus du milieu agricole », qui constituent le principal vivier de ces candidats.

vous pouvez très bien vendre la maison de l’exploitant, voire une partie du bâti agricole à d’autres fins, pour peu qu’il y ait un changement de destination. Ce sera

Elle permettra d’anticiper d’éventuels conflits de voisinage et en facilitera la résolution par les maires ruraux. Lors du congrès de l’Association nationale des élus de la vigne et du vin (Anev), réunie au Palais du Luxembourg le 9 novembre dernier sous la présidence de notre collègue Christian Klinger,

cet article 14, qui vise à créer des zones de transition entre les espaces artificialisés et les espaces agricoles. Le présent amendement

et les nouveaux espaces urbanisés à l’ensemble des communes et non pas seulement à celles qui ont un plan local d’urbanisme. Nous proposons également de renforcer le caractère dérogatoire de la possibilité offerte

où, à titre dérogatoire, la zone de transition serait créée sur l’emprise agricole, nous suggérons d’ouvrir un droit de délaissement au profit du propriétaire du terrain concerné. En effet, la création de la zone de transition peut entraîner une forte perte de valeur du bien. L’équité exige que les propriétaires ruraux ne supportent pas cette perte de valeur. Pour autant, il ne serait pas plus équitable que la commune supporte seule le coût du droit de délaissement. Il est donc proposé

La forte pression de l’urbanisation met en danger les terres agricoles et peut être une source de conflits d’usage entre les agriculteurs et les riverains. Si la protection sanitaire de ces derniers et des utilisateurs des produits phytosanitaires est un impératif, l’agriculture ne doit pas seule en supporter le prix. L’obligation pour les constructeurs de prévoir dans leurs projets une zone de transition répondant aux caractéristiques des zones de non traitement est donc une avancée significative pour la protection du foncier agricole et le maintien des continuités agricoles. par conséquent que les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. Un projet d’urbanisation situé en zone urbaine ou à urbaniser ne peut toutefois se situer simultanément sur l’emprise d’une zone agricole et en zone urbaine ou à urbaniser. Dès lors, la mention « La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture » est nulle et non avenue et la dérogation évoquée hors de propos. On ne saurait accepter que les agriculteurs subissent un recul par rapport aux aménageurs. Le présent amendement a donc

Merci

Si ce constat devait perdurer, voilà qui rendrait impossible la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire des territoires ultramarins fixés par le Président de la République. Il s’agit donc de mettre en place, pour les territoires d’outre mer,

est un des moyens les plus appropriés pour réduire le phénomène des friches. Mais elle est très encadrée. Elle est, du reste, souvent vécue comme une contrainte importante, en raison de l’atteinte qu’elle représente au droit de propriété, qui est un droit constitutionnel.